La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 21 juillet 2022 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Pierre Biarnès, qui fut sénateur représentant les Français établis hors de France de 1989 à 2008. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, qui est en vigueur depuis le 7 juin 2022 dans toute l'Union européenne. Ce règlement européen a pour principal objet d'imposer, dans l'heure, le retrait de « contenus à caractère terroriste » en ligne à tous les fournisseurs de services d'hébergement qui proposent des services dans l'Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal, dans la mesure où ils diffusent des informations au public. Il instaure Il instaure la possibilité pour les autorités nationales d'émettre des injonctions de retrait transfrontalières, exécutoires dans un autre État membre. Enfin, il prévoit que les fournisseurs de services d'hébergement, quelle que soit leur taille, prennent des « mesures spécifiques » pour protéger leurs services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste, dès lors qu'ils sont classés comme étant « exposés » à ces contenus par l'autorité qui en assure la supervision. Ces dispositifs ne sont pas totalement nouveaux en droit français, puisque nous disposons déjà, depuis 2015, de la procédure administrative de retrait prévue à l'article 6-1

La proposition de loi qui nous est soumise est technique ; notre marge de manoeuvre, étroite, est définie par le règlement européen lui-même. Mais la proposition de loi fait relativement consensus sur le fond. Sa constitutionnalité a néanmoins pu susciter un questionnement, au regard de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2020 et relative à la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia. Les circonstances sont toutefois différentes aujourd'hui, compte tenu de l'existence d'une obligation du droit de l'Union. Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord qui conserve les avancées du Sénat. Les autorités compétentes désignées sont celles qui ont déjà l'expérience des procédures administratives de retrait de l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Le suppléant pourra exercer sa mission auprès de la personnalité qualifiée de l'Arcom, lorsque celle-ci exerce ses fonctions dans le cadre de ce même article 6-1. Enfin, et surtout, toutes les injonctions de retrait seront transmises à la personnalité qualifiée, qui pourra ainsi superviser l'ensemble des demandes de retrait concernant les contenus terroristes et saisir le président du tribunal administratif d'une injonction de retrait nationale si celle-ci se révélait non conforme.

le Sénat avait choisi de créer un appel direct devant le Conseil d'État, dans un délai très réduit, pour aboutir rapidement à une décision définitive permettant le cas échéant un rétablissement du contenu supprimé. Cette Cette procédure dérogatoire devant le Conseil d'État n'a pas été retenue par les députés. Dans un esprit de compromis, lors de la commission mixte paritaire, le Sénat a accepté de redonner compétence à la cour administrative d'appel, mais dans des délais réduits : dix jours pour faire appel et un délai maximum d'un mois pour trancher le contentieux. Les membres de la commission mixte paritaire ont également rappelé explicitement l'existence des procédures de référé-suspension et de référé-liberté, cette dernière permettant d'obtenir une décision très rapide en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Le reste des modifications proposées est d'ordre légistique, à l'exception du recours en réformation, remplacé par un recours plus classique en annulation. Les juridictions administratives en effet ne s'estiment pas compétentes pour prendre des décisions à la place de la personnalité qualifiée de l'Arcom ou de l'Arcom

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur-

Grâce à cet accord, la présente proposition de loi permettra de renforcer notre arsenal juridique pour lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. Avec le règlement (TCO), elle constituera un outil décisif dans le combat que nous menons contre le terrorisme en France. Depuis 2017, ce combat a été une priorité du Président de la République et des gouvernements successifs. L'action de l'État s'est concentrée non seulement sur le terrorisme et la radicalisation violente, mais aussi sur les racines du mal. Nous avons renforcé les moyens humains, financiers et juridiques au profit de l'ensemble des services de renseignement, des forces de sécurité et des magistrats qui mènent sans relâche ce combat difficile. Les enjeux de détection, fondamentaux, ont fait l'objet de mesures renforcées, qu'il s'agisse du numéro vert dédié au recueil de signalements- nous devons d'ailleurs rappeler l'importance de ces signalements, car chacun doit se sentir acteur de la lutte antiterroriste -, de l'augmentation des moyens de Pharos, ou encore de la pérennisation de techniques de renseignement innovantes. Ce combat est d'autant plus difficile que les nouvelles technologies du numérique ont facilité la communication transfrontalière et ont contribué à amplifier la circulation de la propagande terroriste. En effet, les actions terroristes sont de plus en plus le fait d'individus qui s'inspirent de messages de propagande émanant des organisations terroristes, incitant au passage à l'acte ou fournissant les tutoriels pour leur réalisation, mais qui ne sont pas pour autant entrés en contact visible ou direct avec des organisations, réseaux ou groupes terroristes. Pour lutter contre ce phénomène, l'Union européenne a adopté en avril 2021, avec le soutien de la France, un règlement relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. Il vise à permettre le retrait des contenus terroristes en ligne en une heure maximum : si les plateformes ne s'acquittent pas de la demande qui leur est faite dans ce délai, elles peuvent se voir infliger des sanctions financières allant jusqu'à 4 % de leur chiffre d'affaires. Ces nouvelles règles s'appliquent depuis le 7 juin 2022, et la présente proposition de loi viendra adapter notre droit pour les mettre en oeuvre. En effet, pour assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, il était indispensable que des autorités indépendantes, chargées d'assurer et de contrôler la légalité du retrait des contenus, soient désignées par chaque État membre. je tiens à saluer votre travail constructif et l'esprit de concorde qui a animé vos débats sur ce sujet si important pour la sécurité des Français. Je remercie le président François-Noël Buffet et la présidente Yaël Braun-Pivet, ainsi que les rapporteurs du texte, MM. André Reichardt et Benjamin Haddad. J'ai également une pensée particulière pour Aude Bono-Vandorme, qui a été à l'initiative de cette proposition À l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, le texte avait été enrichi sur différents aspects. Tout d'abord, la désignation d'un suppléant a été prévue, dans les mêmes conditions que celle de la personnalité qualifiée titulaire, afin de garantir une réponse rapide en cas de sollicitation. Ensuite, en tenant compte des prérogatives dévolues à l'Arcom pour assurer une régulation graduée et effective des contenus, il a été permis à cette instance de mettre en demeure les hébergeurs dès le premier manquement aux obligations administratives concernées, et non aux seuls cas de manquements systématiques ou persistants. En outre, le régime des sanctions a été assoupli pour éviter une double incrimination en cas de non-respect des obligations relatives aux injonctions transfrontalières Enfin, l'Arcom a été dotée de la faculté de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission de suivi des obligations administratives découlant du règlement européen. Le Sénat, quant à lui, a tenu à s'assurer de la transmission systématique à la personnalité qualifiée de l'Arcom des injonctions de retrait au titre de l'article 4 du règlement, afin que la personnalité qualifiée puisse suivre l'ensemble des demandes relatives aux contenus terroristes, sans être limitée aux demandes de retrait formulées au titre de l'article 6-1 de la LCEN et aux injonctions transfrontalières mixte paritaire a également souhaité aligner les peines encourues en cas de non-respect par un fournisseur de services d'hébergement de son obligation d'informer les autorités compétentes d'un « contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie dont il aurait connaissance sur celles qui sont prévues en cas de non-respect de l'injonction de retrait en une heure. En contrepartie, une aggravation des peines a été prévue lorsque la méconnaissance de l'obligation est habituelle. Enfin, au cours de la séance publique, le Sénat a supprimé le mécanisme de double mise en demeure et a souhaité rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de ce règlement. paritaire a permis de valider la procédure juridictionnelle ouverte aux fournisseurs de services d'hébergement et de contenus pour contester les décisions prises par Pharos, par la personnalité qualifiée de l'Arcom ou par cette dernière dans le cadre du règlement européen. Une procédure d'appel devant la cour administrative d'appel a ainsi été prévue, laissant au requérant dix jours pour la saisir, et à la cour un mois

tout en conservant l'esprit initial de ce texte que vous avez largement soutenu. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable au texte issu de la commission mixte paritaire et vous encourage à l'adopter définitivement.

Nous sommes tous conscients de la façon dont internet a facilité la propagande, l'endoctrinement et le recrutement des organisations terroristes. S'il favorise la liberté d'expression, internet sert également à diffuser des idéologies arriérées et barbares, qui s'attaquent à notre modèle de société, à nos valeurs républicaines et à notre sécurité. Il apparaît donc primordial de se doter d'outils juridiques permettant d'entraver et de combattre efficacement l'utilisation d'internet par tous les prédicateurs de haine. Aussi, l'objectif de l'article unique de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne fait largement consensus.

Afin d'aboutir à un texte commun, des ajustements mineurs ont été opérés, portant principalement sur les modalités de recours contre les décisions du président du tribunal administratif.

vous conviendrez que le choix d'une proposition de loi pour transposer les dispositions d'un règlement européen peut nous interpeller ! Cela a été souligné à plusieurs reprises : cette proposition de loi a été rédigée en urgence par les directions centrales des ministères concernés, avant d'être déposée

Avant de conclure, je souhaite saluer la qualité des travaux du rapporteur, M. André Reichardt, malgré les délais contraints. Madame la ministre, mes chers collègues, les discours de haine se propagent et tuent. La menace terroriste demeure l'une des urgences auxquelles notre pays doit répondre. La lutte

Il est en effet de notre responsabilité de prendre toutes les mesures possibles afin de juguler le prosélytisme et de garantir la sécurité physique de nos concitoyens. Vous l'avez compris, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants votera bien évidemment cette proposition de loi.

après une commission mixte paritaire conclusive la semaine passée, je salue aujourd'hui le caractère constructif des travaux ayant conduit à l'adoption de ce texte. L'accord obtenu va nous permettre de lutter avec plus d'efficience contre le partage en ligne des contenus à caractère terroriste, en contraignant les entreprises du Net à supprimer les contenus terroristes en l'espace d'une heure seulement.

Par ailleurs, nous adhérons au compromis trouvé en commission mixte paritaire sur le point non négligeable des procédures de recours. recours. Contrairement au texte adopté par le Sénat, la suite de la procédure d'appel après la première décision du président du tribunal administratif sera portée non pas devant le Conseil d'État, mais devant la cour administrative d'appel, dans des délais brefs. L'appel devra être interjeté dans un délai de dix jours, et la cour administrative d'appel aura alors un mois pour se prononcer. Le choix d'un recours en réformation, plutôt que d'un recours en annulation, nous paraît également plus adapté, compte tenu de la technicité particulière du contentieux à traiter.

qui prévoient la transmission systématique à la personnalité qualifiée de l'Arcom des injonctions nationales de retrait. La personnalité qualifiée pourra ainsi suivre l'ensemble des demandes relatives aux contenus terroristes. Sans cela, il nous aurait paru délicat de garantir la cohérence globale du traitement de ces contenus particulièrement sensibles. En définitive, nous nous félicitions de l'accord obtenu. Je ne doute pas qu'une grande majorité de notre groupe se prononcera en faveur de ce texte, tel qu'il est issu des travaux de la commission Pour finir, le groupe Les Républicains tient à saluer la qualité du travail mené par nos rapporteurs, André Reichardt et Nathalie Goulet,

Nous regrettons ce tour de passe-passe, qui entache la sincérité du processus démocratique. Pour autant, le sujet des contenus terroristes mérite une réponse à la fois pratique, forte et efficace. Nous ne le savons que trop : la haine prolifère en ligne, et nous devons nous doter de l'arsenal le plus efficace possible pour limiter cette propagande terroriste et ces méthodes de recrutement qui ont pour but de nous nuire. Le terrorisme tue, et internet demeure le terreau fertile permettant à la fois la diffusion de certaines idéologies macabres et le recrutement comme le financement des terroristes. Il est essentiel de se doter d'outils de droit freinant cette utilisation Le règlement européen auquel nous devons adapter notre droit est le fruit d'une réflexion sereine. Applicable depuis le 7 juin dernier, il distingue de manière sensée la diffusion de certains de ces contenus à des fins journalistiques, pédagogiques ou artistiques.

La censure de la loi Avia rappelait que la détermination du caractère illicite des contenus à caractère terroriste ne devait pas être soumise à la seule appréciation de l'administration.

» permettant à l'hébergeur d'interdire à un utilisateur de poster du contenu, mais aussi la possibilité d'erreurs techniques inhérentes à des processus automatisés dans la sélection des contenus à supprimer.

Cette différence d'appréciation chez les opérateurs privés pourrait également se retrouver parmi les autorités compétentes équivalentes à l'Arcom. Ce n'est faire offense à aucun de nos voisins européens que de percevoir les nuances dans l'indépendance de ces agences administratives même point de vue sur ce qui caractérise un terroriste. L'aspect transfrontalier des demandes de retrait constitue un sujet majeur, compte tenu de la montée de régimes aux valeurs parfois très éloignées des nôtres au sein même de l'Union européenne. Le règlement auquel nous adaptons aujourd'hui notre droit permet des demandes transfrontalières de retrait de contenus qui pourraient être litigieuses. Comment, sans contrôle d'un juge judiciaire, garantir la liberté d'expression sur notre territoire face à des gouvernements parfois totalitaires, caractérisant de manière caricaturale leurs opposants comme des terroristes ? groupe aurait préféré un meilleur équilibre entre une lutte juste, ferme et efficace contre la dissémination des contenus terroristes sur internet et la protection de la liberté d'expression. Aussi, toutes ces réserves nous empêchent de soutenir pleinement la démarche de la loi

mes chers collègues, le parcours de cette proposition de loi nous laisse très insatisfaits et très critiques, tant sur la méthode que sur les objectifs du Gouvernement. Nous partageons collectivement, sans qu'il soit besoin une nouvelle fois de le la nécessité de lutter contre les propos haineux de toute nature sur internet et les réseaux sociaux. Néanmoins, nous estimons que la technicité de ce dossier, tout comme la nécessité de trouver un juste équilibre entre la régulation des échanges et le respect de la liberté d'expression, aurait justifié de travailler sur un projet déposé par le Gouvernement, à l'occasion d'une navette parlementaire complète. Cette proposition de loi nous prive d'une étude d'impact, de l'avis du Conseil d'État et d'un débat de fond. précédent de la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia, et de sa censure quasi complète par le Conseil constitutionnel aurait dû vous inciter à changer de méthode et à entendre les arguments juridiques forts qui vous ont été opposés. Las ! Nous avons le sentiment que le règlement européen vous donne un prétexte pour nous faire voter ce qui par ailleurs, et à raison, a

de donner aux Sages l'occasion de se prononcer une nouvelle fois sur le régime de protection des libertés individuelles sur les réseaux numériques et de préciser leur jurisprudence sur la liberté qu'ils se donnent de soumettre la législation de l'Union européenne autre de nos réserves porte sur la conformité du règlement, dont la présente proposition se veut la transposition, avec les deux règlements à venir sur les services numériques et sur les marchés numériques, connus sous leurs sigles anglais de DSA () et Dans une formule d'un laconisme absolu, vous nous avez expliqué, madame la ministre, que le règlement 2021/784, adopté le 29 avril 2021, était, je vous cite, « consolidé ». ». Si je comprends bien cet adjectif sibyllin, le Gouvernement estime que les deux règlements à venir ne l'obligeront pas à revoir les dispositions législatives qui seront votées ce jour. De nouveau, j'ai grand-peine à l'admettre, tant les deux règlements DSA et DMA modifient considérablement le statut des hébergeurs de contenus et protègent les auteurs du retrait arbitraire. À tout le moins, une nouvelle fois, notre parlement et les institutions de l'Union européenne ont travaillé en accumulant des dispositifs, sans grande cohérence d'ensemble et sans conférer

pour nous présenter sa politique générale et ses objectifs en vue de la mise en oeuvre des deux nouveaux règlements. Ces règlements auront, dans le champ du numérique, des conséquences sans doute aussi importantes que celles du il eût été de bonne politique que le Gouvernement nous présentât un plan d'action pour leur application en France et qu'il nous informât des moyens nouveaux qu'il pourrait octroyer à l'Arcom et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution Comme le RGPD, ces deux directives auront des conséquences non négligeables sur l'activité d'entreprises étrangères. Sans nul doute, ces dernières-les Gafam, pour ne pas les citer -s'emploieront à les contourner ou à les neutraliser.

Voilà un exemple type de l'endoctrinement terroriste que permet internet et contre lequel nous luttons. Comme notre rapporteur a eu l'occasion de le souligner,

Nous pensons également à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui a imposé aux grandes plateformes numériques une obligation de moyens humains et technologiques proportionnés afin de modérer les contenus ; le tout est placé sous la supervision de l'Arcom. Notre droit doit être outillé ; il le sera encore davantage avec le nouveau dispositif de cette proposition de loi. Il ressortira du règlement européen et de ce texte de quoi continuer à renforcer les prérogatives des pouvoirs publics dans la régulation des contenus en ligne.

! Certes, le cumul de procédures n'est pas idéal. J'ai le sentiment qu'il brouille la lisibilité de la régulation, à laquelle chacun aspire ici. Cela a été beaucoup dit : la méthode législative à laquelle il a été recouru n'était pas la bonne.

Le texte se retrouve examiné à la reprise d'une session parlementaire, nous imposant des délais serrés, entre un projet de loi de veille sanitaire et un autre de mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Bref, nous devons travailler à la hâte : cela n'a rien d'idéal d'idéal ! Chacun s'accordera sur ce point. Les prochaines échéances parlementaires devront mieux tenir compte du temps, du recul et donc de la sérénité qu'impose l'écriture de la loi. Enfin, s'il est question aujourd'hui de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, notre assemblée se préoccupe également du problème des contenus à caractère pornographique, en particulier la mission d'information sur les dérives de l'industrie pornographique.

en adaptant notre législation au règlement européen 2021/784, afin de poser un cadre juridique commun et harmonisé pour l'ensemble des États membres.

parlant, dans ce combat contre les contenus terroristes en ligne ; je pense, par exemple, à la plateforme Pharos. Au cours de la seule année 2021, les enquêteurs de la plateforme dédiée signalement de contenus et comportements illicites en ligne ont formulé pas moins de 10 000 demandes de retrait de publications à caractère terroriste sur les réseaux sociaux. Ces nouvelles dispositions vont permettre de se doter d'outils différents, notre système de défense numérique. Il m'est impossible de voter contre ce texte, n'ignorant pas, en particulier, que la messagerie Telegram a été utilisée par les terroristes du Bataclan. Nous ne pouvons plus nous permettre de telles dérives : il y va de la sécurité de nos concitoyens.

Sous peine de sanctions, il leur revient de détecter et de supprimer le plus rapidement et efficacement possible les contenus de propagande et d'apologie du terrorisme en ligne. Toutefois, la vigilance des des fournisseurs doit être maximale à l'égard de la liberté d'expression et d'information. Le respect de cette liberté fondamentale est le signe d'une bonne santé démocratique. On ne peut négliger cet aspect

J'ai évoqué, lors de la première lecture de ce texte, le récent acte terroriste d'extrême droite commis aux États-Unis, à Buffalo, par un suprématiste blanc. L'auteur a diffusé ses actes en direct sur Twitch. La vidéo dont il est question a été retirée en moins de deux minutes : comme nous l'a rappelé France Culture, « c'est considérablement moins que les 17 minutes qu'il avait fallu à Facebook pour retirer une vidéo similaire, diffusée par le suprématiste blanc autoproclamé qui avait tué 51 personnes dans deux mosquées néo-zélandaises, à Christchurch, en 2019 ces deux minutes ont suffi pour que certains copient les images concernées et les diffusent à leur tour. Le temps réel constitue bel et bien un défi en ce qui concerne le contrôle de la propagation des contenus terroristes en ligne. La proposition de loi que nous examinons en séance a trait à ces enjeux.

de l'étude d'impact et, surtout, de l'avis du Conseil d'État sur la compatibilité du règlement avec notre ordre constitutionnel, un sujet qui a soulevé de nombreuses questions, comme l'a rappelé tout à l'heure notre rapporteur. Peut-être le secrétariat général du Gouvernement, auditionné demain en commission, pourra-t-il nous fournir des explications et répondre à notre souhait qu'il ne soit plus abusé de la procédure législative par voie de proposition de loi.

ou le fournisseur de contenus refuse de se conformer dans l'heure à l'injonction de retrait du contenu, une demande de blocage pourra être adressée par l'autorité administrative au fournisseur d'accès à internet, à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures, conformément à l'article 6-1

et de l'esprit critique et de toute autre initiative permettant de réduire à la fois l'impact des contenus à caractère terroriste en ligne et la vulnérabilité à leur égard. Il ne faut pas sous-estimer l'investissement nécessaire dans le travail social, dans les initiatives de déradicalisation et dans le dialogue avec les communautés touchées,

L'appel interviendra dans un délai de dix jours, devant la cour administrative d'appel, laquelle disposera d'un mois pour statuer. Dans ce cadre, nous soutenons les objectifs des auteurs de cette proposition de loi, qui vise à juguler le plus rapidement possible sur l'espace internet les contenus à caractère terroriste. Je veux particulièrement saluer la qualité du travail des rapporteurs, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, ainsi que de l'ensemble des parlementaires ayant pris part à ces discussions enrichissantes et constructives. Ensemble, il nous faut adresser un signal fort aux entreprises de l'internet, et il nous faut agir d'une seule et même voix, rapidement et efficacement. Sans vouloir paraphraser ce qui a déjà été souligné par mes collègues, il est essentiel de rappeler que ce texte est crucial, pour la sauvegarde de l'ordre public en matière de lutte contre le terrorisme, et, d'autre part, en considération de la situation trouble que l'Europe traverse actuellement. Bien que certaines dispositions de ce règlement figurent d'ores et déjà dans la législation nationale, grâce notamment aux outils ambitieux dont la France s'est dotée ces dernières années, il est essentiel d'en adapter certaines dispositions, afin d'en garantir la conformité. Oui, le terrorisme est une menace qu'il nous faut combattre avec fermeté et sans relâche. la radicalisation et l'incitation à la violence au travers des réseaux sociaux et des plateformes vidéo, ainsi que la diffusion en direct d'attaques, constituent des éléments de plus en plus fréquents dans le cadre des attentats terroristes. Internet en devient indubitablement le principal facilitateur, voire un catalyseur. Les nouvelles technologies sont de précieux atouts pour le progrès humain, pour la diffusion du savoir, pour la coopération internationale, mais aussi pour la résilience de nos sociétés face aux crises ; cependant, elles peuvent également être entravées par les mésusages du numérique. La France prend depuis plusieurs années des mesures ambitieuses pour lutter contre les contenus à caractère terroriste en ligne.

Par ces dispositions, validées par le Conseil constitutionnel, la France a renforcé la lutte contre les « sites miroirs », ainsi que les obligations de moyens des grandes plateformes dans la lutte contre certains contenus illicites, dont la provocation et l'apologie du terrorisme. A également été prévu un pouvoir de sanction du régulateur qu'est l'Arcom.

TCO. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe RDPI soutient pleinement cette proposition de loi, qui met en conformité notre droit national avec le règlement entré en vigueur le 7 juin 2022. juin 2022. Il y va non seulement du respect de nos engagements internationaux et de notre crédibilité auprès de nos partenaires, mais aussi de la sécurité publique dans l'espace cyber. Il est de notre devoir d'accompagner le progrès et l'innovation par un encadrement plus intelligent et plus responsable. Ce qui est proscrit se doit de l'être aussi ! Conformément

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19

nous permettant, après tant de discussions législatives, de sortir définitivement du régime de l'état d'urgence sanitaire et du régime de gestion de la crise sanitaire.

à l'exercer dans de bonnes conditions. Nous avons également fait en sorte que les Français puissent voyager facilement en Europe. Et si l'un des pays membres de l'Union européenne devait ériger des barrières sanitaires à l'entrée de son territoire,

ces deux-là, qui ne sont actionnables qu'en respectant des conditions extrêmement restreintes. Par ailleurs, nous avons veillé à ne pas prendre parti dans le débat d'ordre sanitaire touchant à la réintégration des personnels n'ayant pas voulu se faire vacciner alors qu'ils font l'objet d'une obligation en la matière. Nous avons estimé que ce n'était pas notre rôle que seule une décision médicale, scientifique, pouvait justifier la réintégration de ces personnels. Je rappelle néanmoins qu'ils ont été non pas licenciés, mais seulement suspendus. Par conséquent,

Madame le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, après l'Assemblée nationale hier, il revient désormais au Sénat de se prononcer sur le compromis atteint en commission mixte paritaire sur ce projet de loi. Ce texte aura fait l'objet d'un vif débat, mais la CMP, et c'est heureux, a finalement abouti à un compromis qui entérine la fin de l'état d'urgence sanitaire et du régime d'exception au 31 juillet prochain, tout en maintenant les dispositions minimales et nécessaires pour continuer de protéger les Français. Surtout, ce texte est le résultat d'une méthode, que je souhaite mettre en oeuvre avec vous sur la durée, dans cette situation politique inédite. Cette méthode répond à deux maîtres mots : le dialogue et le compromis, toujours sans compromission. Ce sont toutes les possibilités qu'offre le bicamérisme, le tout au service de la qualité du droit et de la protection de nos concitoyens ; vous savez que j'y suis profondément attaché. Oui, ce texte est une oeuvre collective, alliant les groupes de la majorité et les groupes d'opposition, qui ont répondu à notre appel à ne pas relâcher l'effort face au virus. Je tiens donc à remercier l'ensemble des acteurs de ce compromis.

texte. Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi sur lequel vous allez vous prononcer est un bouclier nécessaire face à une épidémie de covid-19 qui n'a pas dit son dernier mot.

et nous ne pouvons exclure l'apparition de nouveaux variants potentiellement plus préoccupants. En somme, comme je l'ai déjà rappelé, nous devrons toujours et encore être prêts à nous adapter au service de nos concitoyens, notamment des plus fragiles d'entre eux. C'est pour cette raison que ce projet de loi est important et que le texte issu de la commission mixte paritaire est D'une part, ce texte entérine, conformément à l'engagement du Gouvernement et à la situation sanitaire à ce jour, la fin de l'état d'urgence sanitaire et marque un retour bienvenu au droit commun. Ces dispositions devenaient caduques le 1 août prochain, et vous avez choisi de l'écrire explicitement dans la loi. Il ne sera désormais plus possible d'exiger le passe sanitaire pour des actes de la vie courante, comme aller au restaurant. D'autre part, ce texte préserve quelques outils nécessaires, conformément à la rédaction initiale du Gouvernement, pour faire face à une éventuelle recrudescence des cas de covid-19. Des dispositions ciblées sont en effet maintenues pour pouvoir suivre l'évolution de l'épidémie, pour protéger les Français et leur permettre de voyager dans les pays maintenant des restrictions de circulation. En somme, avec ce texte, nous concilions de manière proportionnée la protection des Françaises et des Français avec le respect des libertés individuelles, auxquelles, je le sais, vous êtes tous ici attachés. Surtout, le dialogue entre les deux chambres, notamment le travail exigeant réalisé par la commission des lois du Sénat, a permis d'enrichir ce texte.

également à nous mettre en cohérence avec le règlement européen du 14 juin 2021 relatif au certificat covid numérique de l'Union européenne. Ces dispositions permettront à nos concitoyens de voyager à l'étranger, comme tous les autres Européens, dans le respect des règles établies. De même, la commission mixte paritaire a également permis de confirmer l'apport très important, voté au Sénat, permettant au Gouvernement d'opérer des contrôles sanitaires aux frontières, ainsi qu'entre l'Hexagone et l'outre-mer. Vous le savez, cet outil est essentiel pour nous permettre de réagir rapidement en cas d'apparition d'un variant préoccupant ou à risque avéré. J'avais dit, après la suppression de cet article, que je voulais me battre pour le réintégrer. Je me félicite donc du fait que vous ayez permis son retour. Je remercie de nouveau Philippe Bas et les groupes de gauche, de droite et du centre qui ont largement voté cette disposition. En revanche, vous avez souhaité que cet article soit limité aux tests de dépistage de la covid-19, alors que le projet initial du Gouvernement visait aussi les preuves de vaccination ou de rétablissement. L'objectif était de pouvoir protéger de manière plus efficace nos concitoyens en disposant d'une boîte à outils qui nous permette de nous adapter à toutes les situations, en cohérence avec les choix de nos voisins ou de pays plus lointains. Toutefois, le compromis parlementaire s'est établi ainsi. Par ailleurs, la question de la réintégration des professionnels soumis à l'obligation vaccinale a également fait l'objet, à mon sens, d'un traitement équilibré et responsable. Je soutiens le consensus issu de la commission mixte paritaire, qui s'appuie, comme je l'ai toujours souhaité, sur l'avis des scientifiques et de la Haute Autorité de santé. Enfin, le Parlement a souhaité que le Gouvernement présente un rapport exposant le cadre juridique existant pour lutter contre les pandémies et les évolutions possibles pour limiter le recours aux régimes d'exception. Je répondrai à cette demande et je m'attacherai à ce que ce rapport puisse au mieux éclairer et enrichir le travail de contrôle et d'évaluation du Parlement. Mesdames, messieurs les sénateurs, je terminerai en un mot : le texte sur lequel vous allez vous prononcer est le fruit d'un travail parlementaire consensuel et exigeant, que le Gouvernement respecte. C'est aussi et surtout un outil profondément nécessaire de protection de la santé des Français à laquelle, par-delà les différences politiques, nous sommes tous attachés. Nous passons

avec l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire d'un treizième projet de loi sanitaire. Comme ce fut le cas par le passé, ce texte comprend un certain nombre de dispositions destinées à doter les pouvoirs publics d'outils servant à accompagner

ce projet de loi se caractérise par un contexte particulier, puisque les régimes dérogatoires mis en place ces deux dernières années arriveront à leur terme ce dimanche. La question était donc de savoir quels outils nous souhaitions conserver temporairement. Or, tandis que la septième vague de l'épidémie de covid-19 est toujours en cours, le Gouvernement a souhaité prolonger deux dispositifs : les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid et le mécanisme permettant l'instauration de contrôles sanitaires

je tiens à saluer le travail, afin de remanier en profondeur le projet de loi dans le sens d'une plus grande proportionnalité, de la responsabilité et de la clarté. Nous avons tout d'abord décidé d'inclure explicitement dans la loi l'abrogation des différents dispositifs dérogatoires du droit commun qui s'étaient accumulés dans les textes depuis mars 2020. À l'avenir, réactiver un régime d'exception nécessitera de remettre entièrement l'ouvrage sur le métier devant le Parlement. ensuite voté l'ajustement du dispositif juridique concernant le système d'information, qui permettra de conserver l'accès des Français au certificat covid numérique de l'Union européenne entre janvier et juin 2023,

à l'obligation vaccinale, nous avons souhaité offrir une perspective de réintégration aux personnes suspendues, qui ont nécessairement vocation à être réintégrées. La décision de cette réintégration, comme l'a souligné notre rapporteur, relevait jusqu'ici du seul Gouvernement : le Sénat a fait en sorte que ce soit la Haute Autorité de santé qui en décide le moment venu.

En effet, il est question non plus de donner carte blanche au Gouvernement pour instaurer des contrôles sanitaires généralisés, mais plutôt de limiter cette possibilité aux voyageurs en provenance de pays où l'apparition de nouveaux variants pourrait susciter des risques sanitaires particulièrement graves. En cas d'activation de ces dispositifs, les voyageurs concernés devront fournir un test virologique négatif.

Enfin, en cohérence avec ses positions sur les textes sanitaires précédents, le Sénat avait prévu que le Gouvernement soit tenu de demander au législateur la prolongation de toutes ces mesures au-delà d'une durée initiale limitée.

Certes, il limite la présentation d'un certificat de voyage aux personnes venant de l'étranger ou à toute personne souhaitant se rendre dans les collectivités ultramarines, mais il maintient cette obligation dès l'âge de 12 ans et ne rend pas les tests gratuits pour tous. Notre groupe reste persuadé que toute modification significative des libertés, telle que celle d'aller et venir, doit se faire de manière non seulement concertée, mais surtout éclairée et précise. Éclairée, en ce que le Parlement doit bénéficier des mêmes informations que l'exécutif. Il est regrettable, pour ne pas dire plus, que nous ne soyons pas destinataires de manière concomitante au Gouvernement ou au Président de la République des travaux du Conseil scientifique.

Le refus du Gouvernement d'inscrire des seuils ne nous étonne plus : les seuls seuils d'alerte qu'il s'était lui-même imposés depuis quelques mois n'ont eu aucun impact sur sa propre gestion de la crise ... Quant à la saturation du système de santé, je ne vous

Bien avant que le Gouvernement n'engage la discussion sur la troisième dose, nous l'avions alerté sur les disparités vaccinales en lui demandant de s'attacher à comprendre et combattre de tels déséquilibres. Pourtant, alors qu'à peine plus d'un quart des plus de 75 ans ont un schéma vaccinal complet, à savoir deux doses et deux rappels, le Gouvernement détourne le regard des plus fragiles, des plus précaires, des plus éloignés de l'épicentre de notre vie sociale.

la qualité de l'air. Mais il n'y a toujours aucun plan ni aucune mesure solide sur l'air des lieux fermés, comme les écoles, dont la sécurisation devrait être votre priorité. Nous attendions des mesures fortes dès maintenant pour aller vers les populations non vaccinées, des mesures claires sur le prix des masques efficaces, comme les FFP2, et sur la gratuité des tests de dépistage, particulièrement essentielle pour ne pas faire des Ultramarins et des Français de l'étranger des citoyens de seconde zone. des rappels forts de l'importance des gestes barrières, pour ne pas transformer le vaccin ou le passe sanitaire en un outil à effets pervers. Nous souhaitions des discussions éclairées sur l'avancée des données scientifiques quant à l'efficacité éventuelle des vaccins sur de nouveaux variants ou sur la nécessité de conserver ou non les données en jeu à l'article 1. Nous demandions des actes et un accompagnement financier sur la qualité de l'air dans nos écoles, maintes fois repoussés et désormais promis par le Président de la République. Enfin, nous proposions un dialogue réel sur les dangers connus, les dangers prévisibles et les retours d'expérience de la gestion de ces deux dernières années par votre gouvernement.

Ainsi, le Gouvernement ne pourra plus réactiver simplement un passe sanitaire ou vaccinal, ni confiner la population sans repasser devant le Parlement avec un nouveau texte et de nouvelles mesures, qui seraient alors débattues et votées. C'est ce qu'implique l'abrogation complète des dispositifs exceptionnels de lutte contre la pandémie. Cette mesure emporte notre approbation, tout comme l'instauration d'un mécanisme de protection sanitaire aux frontières si un nouveau variant très dangereux apparaît. Un test pourrait alors être exigé pour l'accès au territoire. Nous n'y sommes pas défavorables non plus, à un bémol près l'applicabilité de cette mesure aux jeunes de 12 à 18 ans. Nous avions proposé, en séance publique, que le certificat sanitaire de voyage ne soit pas applicable pour les 12-18 ans,

Par ailleurs, nous nous interrogeons fortement sur le sort qui serait réservé à nos concitoyens ultramarins si ce certificat sanitaire de voyage devait entrer en vigueur.

en ce qui concerne la réintégration des personnels non vaccinés, notre rapporteur a décidé d'évacuer la question en renvoyant la décision à la Haute Autorité de santé, que le Parlement pourra saisir. À elle de décider de la réintégration de ces personnels, s'il est constaté que l'obligation vaccinale n'est plus médicalement médicalement justifiée. Pour notre part, nous pensons que ces personnels devraient immédiatement être réintégrés : comme chacun le sait, le vaccin n'empêche pas d'être porteur du virus, et c'est d'ailleurs bien la logique que vous avez adoptée, mes chers collègues, en instaurant un certificat sanitaire de voyage nécessitant uniquement un test négatif et non un schéma vaccinal complet. De plus, si ces personnels avaient été suspendus, ce à quoi nous étions fermement opposés, c'était pour protéger les plus vulnérables au service desquels ils étaient amenés à travailler et non pour les protéger eux-mêmes d'un risque de contamination. Aujourd'hui, on nous présente le schéma inverse : ces personnels devraient continuer d'être suspendus, car leur non-vaccination les exposerait à développer une forme de covid dangereuse pour leur propre santé

Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis, si la situation sanitaire semble stable et sous contrôle, et bien que les nouvelles admissions à l'hôpital tendent à augmenter légèrement, ces indicateurs doivent être mis en perspective avec les fragilités que connaît le système de soins. Que Que propose le Gouvernement en la matière ? Rien, sinon vivre avec le virus. Ce dernier ne devrait-il pas nous pousser à engager une réforme d'ampleur face à l'état d'urgence de nos hôpitaux qui, lui, n'a jamais cessé, et face à la casse généralisée et désormais totalement assumée de notre système public hospitalier ? Monsieur le ministre, que vous inspirent les quelque 150 services d'urgences qui ont manifesté leur détresse depuis la fin du mois de mai dernier ? Que vous inspire l'hémorragie de fermetures de lits d'hôpitaux ? Il s'agit là de questions

Comme chacun d'entre vous, j'ai pris connaissance du dernier avis du Conseil scientifique en date du 19 juillet dernier, qui insiste sur la nécessité

nous examinons aujourd'hui le premier texte de la législature issu d'un accord rapide entre députés et sénateurs, et ce dès la première lecture. Le texte a été adopté hier par l'Assemblée nationale.

Toutefois, je tiens à exprimer de nouveau ici mes regrets quant à la voie qui a été choisie. Un contrôle sanitaire pourra être instauré aux frontières de l'Hexagone en cas de résurgence d'un variant du covid ou de saturation des hôpitaux outre-mer, mais seul le test fera foi. Nous sommes nombreux à regretter la suppression de la preuve vaccinale et du certificat de rétablissement. Le débat a laissé le champ libre aux antivax, alors que les faits sont clairs : en plus de protéger la personne concernée, le vaccin, je le répète, limite la circulation virale et en réduit la contagiosité.

? Le problème tient aussi au message adressé. Alors que les vaccins anti-covid ont sauvé des millions de vies, ils seraient aujourd'hui devenus inutiles pour lutter contre la diffusion d'un variant dangereux, avant même que les autorités médicales ne s'expriment

Sur le fond, cet article ne change rien au droit actuel, hormis l'automaticité de la réintroduction des soignants non vaccinés, dès que la Haute Autorité de santé aura jugé l'épidémie éteinte. Après deux avis similaires rendus par le conseil scientifique et l'Académie de médecine, la HAS a tranché la semaine dernière. Elle s'est déclarée de nouveau favorable au maintien de l'obligation vaccinale contre le covid-19 pour les personnels des établissements de santé et médico-sociaux, compte tenu des « incertitudes sur l'évolution de l'épidémie » et de l'« efficacité d'un schéma vaccinal complet à réduire le risque d'être infecté et de transmettre la maladie ». Toutes les autorités scientifiques s'accordent sur ce sujet. Il est donc regrettable de voir nos assemblées parlementaires jouer sur une forme d'ambiguïté, qui aurait pu mener,

été repris par la commission mixte paritaire. Le Parlement devra ainsi autoriser ce contrôle aux frontières, s'il est prolongé au-delà de deux mois. Le changement de titre, souhaité par notre rapporteur, offre par ailleurs une clarification bienvenue. Les réseaux antivax et antipasse se sont réactivés à l'approche de l'examen de ce projet de loi, diffusant des messages mensongers sur une possible prolongation de l'état d'urgence. La nouvelle dénomination permet ainsi d'établir clairement la fin des régimes d'exception. Le plus dur semblant être derrière nous, il paraît logique de revenir à des procédures plus classiques pour un virus lui-même plus classique. Nous devons continuer, collectivement, à lutter contre la désinformation, en prenant des décisions fondées sur les données scientifiques. Le Gouvernement a également un rôle majeur à jouer dans la communication des mesures efficaces de lutte contre le covid : gestes barrières, aération des espaces clos, politique vaccinale. À ce jour, je le rappelle, moins de 30 % des plus de 60 ans ont reçu leur deuxième dose de rappel. Mais une meilleure communication est aussi attendue du corps médical s'agissant des nouveaux traitements disponibles, efficaces dans certaines indications. Il y va de la responsabilité de chacun.

nous le savons, l'épidémie n'est pas encore derrière nous, 1 300 personnes étant aujourd'hui hospitalisées en soins critiques. Par ailleurs, nous ne sommes pas à l'abri de l'apparition d'un nouveau variant plus dangereux, qui viendrait accroître la tension

SI-DEP, pilier de la lutte contre l'épidémie, est indispensable. La date finalement retenue du 30 juin 2023 me semble toutefois bien lointaine. Il eût été judicieux d'introduire une clause de revoyure

En cas de mise en place du dispositif, seules les personnes disposant d'un schéma vaccinal complet ou d'un certificat de rétablissement pourraient prétendre à la gratuité des tests. Or ce certificat possède une durée de validité de six mois. De ce fait, le test sera payant passé ce délai. Je vois dans une telle situation une réelle inégalité. En octobre 2021, la Défenseure des droits alertait déjà sur le caractère discriminatoire du non-remboursement des tests pour une partie de la population. La solution est pourtant simple : la gratuité des tests pour toutes et tous, vaccinés, non vaccinés et rétablis de la covid. Si ce texte incarne notre relative adaptation à l'épidémie, il ne permettra pas à l'ensemble de la population de vivre de façon égale avec ce virus. C'est pour cette raison que je m'abstiendrai. Ce n'est

de détermination et de courage. J'ai entendu vos propos, monsieur le ministre. Votre gouvernement s'est présenté avec un texte que l'on pourrait qualifier de « minimal

C'est ainsi que le régime d'exception a été abrogé. Toutefois, de manière inquiétante, le rôle du Parlement, et singulièrement du Sénat, s'en est trouvé dévalorisé.

Nous avons vu le vaccin retiré du passe sanitaire, alors que, depuis deux ans, nous plaidons sans relâche auprès de nos compatriotes pour qu'ils soient vaccinés,

et dangereux, voire inconstitutionnel. Malgré cela, M. le rapporteur et l'ensemble de la majorité du Sénat, que l'on a connus plus exigeants sur ces sujets, ont accepté de passer par-dessus ces difficultés

effet, les missions de santé, c'est-à-dire les obligations de l'État pour faire face aux crises sanitaires, déjà connues ou potentielles, sont une responsabilité première de l'État, à laquelle le Parlement doit apporter toute son attention.

de ce qui a fonctionné et de ce qui est reproductible parmi les mesures de précaution et de prévention, qui sont de la nature même du code de la santé publique,

est honorable pour tous les participants. Nous constatons que les votes ont évolué positivement à l'Assemblée nationale

Gouvernement réfléchira à une évolution, éventuellement à une levée de l'obligation vaccinale, il devra le faire de façon différenciée, car la situation des soignants « directs », si j'ose dire, c'est-à-dire des agents en contact avec les malades et les

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Fort heureusement, ces contaminations n'ont plus les conséquences dramatiques massives d'il y a deux ans. Les hospitalisations ne submergent plus notre système de santé, bien que le virus continue de tuer. La couverture vaccinale de notre pays permet de faire face à l'afflux de patients qui ont besoin de soins. Dans ces conditions, le Gouvernement n'a pas souhaité proroger l'état d'urgence sanitaire après le 31 juillet prochain. Il a proposé au Parlement de prolonger certaines mesures de veille et de surveillance de l'épidémie. Après un examen rapide par les deux chambres du Parlement, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur ce texte, reprenant bon nombre des ajouts et modifications adoptés par le Sénat. Afin d'envoyer un message clair à nos concitoyens, notre commission a fait le choix d'abroger les dispositions de l'état d'urgence sanitaire, qui étaient vouées à devenir caduques le 31 juillet. Les traitements de données nécessaires à la surveillance de l'épidémie sont prorogés de quelques mois. Bon nombre de situations exigent toutefois le recueil du consentement des personnes concernées. Le Sénat a par ailleurs rétabli l'article 2 du projet de loi, qui prévoit la possibilité de contrôler les déplacements entre les outre-mer et la métropole, ainsi qu'entre l'étranger et le territoire national. Cet article avait été rejeté par l'Assemblée nationale, bien que les amendements de suppression n'eussent pas été adoptés.

combien la vaccination est utile et importante. Nous aurions souhaité qu'un justificatif de vaccination ou qu'un certificat de rétablissement, le cas échéant, Une autre disposition majeure du texte concerne la réintégration des soignants non vaccinés. Aucune mesure du projet de loi initial ne modifiait le régime actuel : cette réintégration était possible par décret du Gouvernement pris après avis de la Haute Autorité de santé. La commission des lois a souhaité que la HAS devienne décisionnaire sur cette question. Nous le regrettons, car il nous semble qu'il y va d'une décision éminemment politique, qui aurait dû rester entre les mains du Gouvernement. Il faut souligner en effet que les soignants, dans leur très grande majorité, ont fait le choix de la vaccination, parce qu'ils ont à coeur de protéger les patients et parce qu'ils ont confiance dans la science, dont ils sont Si actuellement le virus n'est plus aussi dangereux qu'auparavant, si les contraintes s'allègent, si la vie des Français se dirige de plus en plus vers un retour à la normale, c'est bien grâce à ceux qui ont fait le choix de se vacciner et non grâce à ceux qui ont refusé

Quoique ce projet de loi contienne des mesures nécessaires, certaines de ses dispositions ne satisfont pas pleinement l'ensemble de notre groupe. Aussi chacun d'entre nous votera-t-il en fonction de ses convictions. C'est beau